voter contre. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

tenues de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus de la covid 19, tel qu’il résulte des articles 5 et 6 de la loi n° 2020 473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Ces équipements de protection individuelle sont nécessaires aux professionnels de santé, pour des raisons de sécurité sanitaire.

entreprises étrangères dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 85 000 euros pour leurs opérations réalisées en France. Pour qu’elles en bénéficient, le chiffre d’affaires européen de ces très petites entreprises (TPE) doit en outre être inférieur à 100 000 euros. Cependant, il n’existe pas d’obligation d’identification en France. L’ensemble des formalités sont en effet réalisées dans l’État de résidence de l’entreprise étrangère, qui transmet ensuite les informations à la France. Afin de limiter le coût du risque de fraude qui en découle, nous proposons de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui qui a été retenu en loi de finances 2024. Enfin, il s’agirait aussi d’une véritable mesure d’économie pour les finances publiques, car il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes de

cumule harmonisation, simplification et contribution budgétaire sans trop pénaliser les entreprises concernées.

M. Thierry Cozic. Les opérations de bail réel solidaire – les fameux BRS – portant sur les logements anciens sont soumises à la perception de droits taux plein une première fois lors de l’acquisition réalisée par l’organisme de foncier solidaire, puis une seconde fois lorsque les droits sur le bâti sont cédés aux ménages. afin d’éviter cette double peine, il est proposé de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les organismes de foncier solidaire au droit fixe de 125 euros, la cession des droits aux ménages restant quant à elles soumise aux droits d’enregistrement, selon les règles de droit commun. Quel est l’avis de la commission

l’habitation pour les logements locatifs sociaux situés outre mer a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité (SLS). Le taux applicable est au maximum de 2,5 % sur les loyers

Comme cela a été très justement rappelé, en Guyane, les agriculteurs ne parviennent pas à accéder au foncier, alors même que ce territoire couvre 8,4 millions d’hectares. De fait, 90 % des terres sont encore considérées comme appartenant à l’État du fait de l’application de la doctrine coloniale de la. Depuis Depuis 2016, le schéma d’aménagement régional prévoit 75 000 hectares de surface agricole utile. Pourtant, dans le cadre de l’accord conclu après le mouvement social de mars et avril 2017, l’État n’a cédé que 20 000 hectares à la amendement vise simplement à relever les défis de la souveraineté alimentaire et de l’organisation de la filière agricole. Plus de deux tiers des jeunes sortis du lycée agricole ne parviennent pas à s’installer, faute d’accès au foncier. L’amendement tend à ce que l’État transfère à la Safer entre 125 000 et

Or l’inventaire des terrains cessibles, réalisé par la Safer avec l’aide de la Fédération nationale des Safer (FNSafer) et des services de l’État en Guyane, est maintenant complet. L’État doit donc attribuer au plus vite les 20 000 hectares prévus afin que la Safer de Guyane puisse réellement œuvrer au développement agricole du territoire.

entraîne obligatoirement, et pour la durée de l’accord, une baisse effective du prix pour le consommateur. Les observatoires des prix, des marges et des revenus seront garants de ce blocage des prix. La parole

notamment en Martinique. Le coût de la vie est particulièrement élevé dans ces territoires. Les produits de première nécessité y sont bien plus chers qu’en métropole, ce qui pèse fortement sur le pouvoir d’achat des habitants. Deuxièmement, la réduction de TVA permettra d’alléger immédiatement ce fardeau.

permettront un contrôle rigoureux des prix. Pour garantir que la baisse décidée bénéficie réellement aux consommateurs, l’observatoire des prix, des marges et des revenus surveillera l’évolution des prix et signalera toute hausse injustifiée. Cette transparence assurera le respect de l’accord et protégera les consommateurs.

du droit de partage de 2,5 % pour les immeubles situés dans les territoires ultramarins concernés par le dispositif dérogatoire de sortie de l’indivision.

L’obligation de réception des factures électroniques par toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, est ainsi fixée au 1 septembre 2026. L’obligation de facturation électronique et de transmission des données pour les opérations de vente est également

il apparaît que les facturations mensuelles du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) ne sont pas traitées par les spécifications externes de la facturation électronique en B to B qui définissent les circuits de facturation. La liste des plateformes partenaires retenues dans le cadre de la première étape de la procédure d’immatriculation vient d’être publiée officiellement.

Fragilisée par la crise, la société française Corsair en a bénéficié, dans le cadre d’un plan de restructuration. Celui ci reposait en partie sur le soutien financier de l’État, notamment au travers de l’aide fiscale. en raison de la prolongation des effets de la crise et de l’augmentation significative du prix des carburants, ce plan de restructuration n’a pas permis à la compagnie d’achever le redressement de sa situation financière. amendement vise donc à rétablir, sous certaines conditions, et avec l’approbation de la Commission européenne, la mesure dérogatoire permettant à Corsair de bénéficier du crédit d’impôt précité entre le 1 janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

En 2023, la CTM a soutenu 1 300 entreprises, 50 associations sportives et 120 associations culturelles ; elle a ainsi fourni des prestations à des milliers de bénéficiaires.

Ces restrictions affecteront inévitablement le service public et limiteront l’investissement public local, dont la CTM assure les deux tiers. Les

sur une liste de produits de première nécessité, en concertation avec l’ensemble des acteurs intégrés dans la chaîne logistique et d’approvisionnement des biens de consommation. Cela assurera

Depuis 2017, l’exécutif a vidé les caisses de l’État en multipliant les avantages fiscaux en faveur des grandes entreprises. Or, aujourd’hui, il semble enfin prêt à reconnaître la nécessité de les faire contribuer davantage.

Cette temporalité risque d’avoir un effet pervers : certaines entreprises pourraient choisir de reporter des opérations ou de limiter artificiellement leurs profits sur la période concernée, afin d’échapper à la taxe.

En vous décidant enfin à instaurer une taxe sur les profits des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros, vous exécutez un très léger pas de côté par rapport à votre fiscal des grandes entreprises de ce pays, pays, lesquelles semblent plutôt bien se porter : elles ont redistribué 150 milliards d’euros de dividendes l’an passé, un record. Il faut noter que cet article ressemble fortement, au moins dans l’idée, à la taxation des superprofits défendue par notre groupe depuis la crise sanitaire.

il instaure une contribution exceptionnelle temporaire sur les bénéfices des grandes entreprises. L’impôt sur les sociétés fait partie des impôts principaux, que nous examinons avec les recettes dans cette première partie,

à hauteur de 56,2 milliards d’euros pour 2025. Cette contribution exceptionnelle avait été mise en œuvre dans les années notamment en 1974 à la suite du premier choc pétrolier de 1973, et à plusieurs reprises, jusqu’en 2017,

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

! – pour les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros.